d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. L'ordre du jour appelle, à la demande du groupe Union Centriste, la discussion de la proposition de loi visant à créer un droit à l'erreur des collectivités locales dans leurs relations avec les administrations et les organismes de sécurité sociale, présentée par M. Hervé Maurey, Mme Sylvie Vermeillet et plusieurs de leurs collègues Dans la discussion générale, la parole est à M. Hervé Maurey, auteur de la proposition de loi. Monsieur

pour les particuliers et les entreprises dans leurs relations avec les administrations. Nous nous en réjouissons. Lors de l'examen de ce texte, le Sénat, sur l'initiative de notre collègue Sylvie Vermeillet, avait étendu cette disposition aux collectivités locales et à leurs groupements, contre l'avis du Gouvernement.

Ce point de désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat a d'ailleurs été l'une des causes de l'échec de la commission mixte paritaire sur ce texte, qui n'a donc pas repris le dispositif. Attaché à la reconnaissance de ce droit pour les collectivités, j'ai souhaité, avec Sylvie Vermeillet, reprendre ce dispositif dans une proposition de loi, en le limitant aux communes et à leurs groupements, qui sont sans doute les collectivités locales les plus concernées.

Je suis donc très heureux que cette proposition de loi soit aujourd'hui inscrite à l'ordre du jour de la Haute Assemblée à la demande du groupe Union Centriste, que je remercie. Je remercie également le rapporteur, Philippe Bonnecarrère, qui, comme toujours, a travaillé avec beaucoup de rigueur et d'intelligence sur ce texte ... C'est très vrai Je remercie évidemment le président de la commission des lois, l'excellent Philippe Bas, et l'ensemble de ses membres, qui ont unanimement voté ce texte. L'application du droit à l'erreur aux collectivités locales me paraît en effet pleinement justifiée. Les collectivités locales sont, dans certains cas, des usagers des administrations dans les mêmes conditions que les particuliers et les entreprises. Elles s'acquittent ainsi de cotisations sociales et reversent le prélèvement à la source en tant qu'employeur. Dans certains cas, elles peuvent être assujetties à la TVA dans le cadre de certaines de leurs compétences- fourniture d'eau, transport de personnes, déchets, Le risque pour une commune de commettre des erreurs s'est accru au cours des années avec la multiplication des normes et la complexification des procédures administratives. Ce risque est particulièrement réel pour les petites communes, qui disposent non pas de services juridiques aguerris, mais simplement, quelques heures par semaine, d'une secrétaire de mairie qui, quelles que soient ses compétences et son implication généralement exemplaires, ne peut pas, tant sa tâche est diverse et lourde, connaître l'ensemble des règles administratives complexes et changeantes. En outre, sous l'effet des réorganisations successives des services de l'État, se traduisant par des baisses d'effectifs, les communes ne bénéficient plus dans les mêmes conditions de leur appui juridique et de leurs conseils. Or une erreur peut avoir des conséquences particulièrement préjudiciables pour une collectivité locale, notamment d'un point de vue financier. Certaines erreurs peuvent même conduire celle-ci ainsi que les élus à voir leur responsabilité engagée. On sait à quel point ce sujet est source d'angoisse pour les élus. Les récents travaux du Sénat sur l'exercice du mandat d'élu local l'ont rappelé. Si nous pouvons espérer que le rescrit administratif créé par la loi du 27 décembre 2019 sera utile, il y a tout lieu de penser qu'il ne sera pas suffisant compte tenu du nombre de décisions prises par les collectivités et de son caractère peu contraignant pour le préfet. Il faut Il faut donc offrir aux communes comme aux citoyens et aux entreprises une seconde chance en cas d'erreur commise de bonne foi. Tel est l'objectif de ce texte, qui constituera donc un « nouveau » droit pour les communes et confirmera la volonté de la Haute Assemblée de répondre aux attentes de nos collectivités locales. La parole

vous toutes et vous tous, mes chers collègues, qui portez sans faille la cause des communes et des collectivités territoriales. Je remercie en particulier Hervé Maurey, sans qui cette proposition de loi n'aurait probablement pas vu le jour. C'est lui qui a pensé que mon amendement initial devait devenir un texte de loi. Bonne idée, en effet ! Je témoigne de ma chance d'avoir pu bénéficier de sa belle expérience. Je remercie également le groupe Union Centriste de nous faire confiance en nous permettant de vous présenter nos travaux. Merci aux membres de la commission des lois, à son président et, bien sûr, à notre excellent rapporteur Philippe Bonnecarrère, qui a ciselé la proposition de loi avec l'exigence et la finesse que nous lui reconnaissons tous. Ainsi, monsieur le rapporteur, vous avez su valablement faire évoluer ma propre conception du droit à l'erreur en démontrant qu'il était nécessaire d'en préciser le champ d'application et d'éluder l'ambiguïté de la collectivité tantôt puissance publique tantôt usager. Monsieur le secrétaire d'État, dans le prolongement de l'intervention du président Maurey, je voudrais dire que, nul doute, les collectivités méritent le même droit à l'erreur que l'ensemble des bénéficiaires de la loi Essoc. Ma courte intervention voudrait appeler votre attention sur le fait qu'elles en ont besoin. Premièrement, comment la fonction publique territoriale, avec ses 2 millions d'agents, ne serait-elle pas légitime dans ses relations avec l'Urssaf ? L'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale prévoit bien le contrôle des employeurs privés et publics Les collectivités sont contrôlées comme le privé ! Il n'y a jamais que 75 550 comptes d'administrations et de collectivités territoriales dans les Urssaf, avec, en moyenne, un redressement dans les deux tiers des contrôles des exemples dans le Nord. En avril 2019, la commune de Beuzeville a dû payer 202 270 euros à l'Urssaf pour avoir appliqué une exonération de cotisations sociales à l'ensemble du personnel d'aide à domicile

En 2018, en Bretagne, sur 71 collectivités contrôlées, 99 653 euros de redressements ont été prononcés, dont 80 % au bénéfice de l'Urssaf. Partout, les erreurs existent. Toutes les collectivités sont donc légitimes à bénéficier du droit à l'erreur.

Et la TVA, ce sont bien des tracas ! Comment s'y retrouver dans les exclusions de base d'imposition, les franchises, les biens immobiliers, les livraisons à soi-même, les prestations entre collectivités, de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée) ? Comment n'y aurait-il pas d'erreurs ? Pourquoi n'y aurait-il donc pas de droit à l'erreur ? Le tribunal d'Amiens a donné raison à une commune qui n'avait pas appliqué la TVA à une vente de terrain à une société d'HLM pour un montant de 359 450 euros. L'administration fiscale l'exigeait pourtant très sérieusement Monsieur le secrétaire d'État, puisque la loi Essoc s'articule autour de deux piliers- faire confiance et faire simple -, puisque la loi Engagement et proximité, s'en inspirant, a étendu la procédure de rescrit aux collectivités, puisque les premiers résultats vous ont conduit à créer le site simplifions@modernisation.gouv.fr afin de permettre aux contribuables d'exprimer leurs difficultés ou de faire part de leurs solutions, mon seul message, à cet instant, est de souscrire à tout cela, d'inscrire les collectivités dans le partenariat et la simplification. Je dirais même dans la contribution aux solutions, car, en matière de normes excessives, elles ont beaucoup à dire et à témoigner. Notre interaction vaut tellement mieux que nos confrontations ! Parce que c'est en fait l'ensemble du pays qui revendique notre synergie, l'État doit accorder le droit à l'erreur aux collectivités ; il peut même imaginer que les collectivités vont l'aider à corriger des erreurs. corriger des erreurs. À quelques mois des municipales, vous pourriez envoyer un signal : que le droit à l'erreur soit, de fait, le droit au meilleur !

je ne suis pas sûr de pouvoir immédiatement illustrer le droit au meilleur réclamé par notre collègue Sylvie Vermeillet il y a quelques secondes. Ni plus ni moins et pas d'impunité C'est ainsi que je résumerai l'intention d'Hervé Maurey et de Sylvie Vermeillet, les auteurs de la proposition de loi qui nous est soumise. En demandant que les collectivités, lorsqu'elles sont usagères, bénéficient du droit général à la régularisation en cas d'erreur existant au profit des particuliers et des entreprises, nos collègues souhaitent que les collectivités n'aient ni plus ni moins de droits que les particuliers ou les entreprises. Ils demandent non pas une dérogation, mais le régime commun ; ils ne nous soumettent pas un texte d'impunité ou un texte de faveur. La création d'un droit à l'erreur, plus exactement d'un droit général à régularisation en cas d'erreur, a été la mesure emblématique d'une loi de 2018, la loi Essoc. L'idée du droit à régularisation, sauf mauvaise foi ou fraude, a trouvé sa place dans un code- il en existe pas mal -, à savoir le code des relations entre le public et l'administration, le CRPA. Mme Vermeillet avait demandé à l'époque, par voie d'amendement, l'extension du droit à régularisation aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Le Sénat y avait été favorable.

Vous avez donc, chers collègues, dès 2018, approuvé cette extension, et notre commission des lois, la semaine dernière, à l'unanimité, a approuvé l'objectif porté par les auteurs de la L'intérêt principal du débat de cet après-midi serait de vous convaincre, monsieur le secrétaire d'État. Si nous y parvenons, il n'est pas interdit de penser que vous saurez convaincre l'Assemblée nationale. Vous le savez tous, chers collègues, le Gouvernement veut se réconcilier avec les collectivités, dit-on, trouver la voie d'une confiance réciproque, monsieur Collombat, et supprimer les irritants. Nos collègues, monsieur le secrétaire d'État, vous proposent de supprimer un irritant

Tout en respectant la volonté de nos collègues, nous avons essayé de réécrire le texte en tenant compte de vos réserves et de vos critiques. Comment ? Premièrement, vous nous avez dit, en 2018,

ajoutiez-vous, ce droit a été inséré dans le code des relations entre le public et l'administration. L'étendre au bénéfice d'autres administrations risquerait de diluer l'objectif clairement affiché sur cette mesure centrale du projet de loi, qui s'adresse aux usagers dans leurs relations avec toutes les administrations. Soit, monsieur le secrétaire d'État, ne diluons pas Nous avons donc supprimé toute référence au CRPA. Nous proposons la création d'un droit à l'erreur autonome dans le seul code général des collectivités territoriales, là où il doit finalement être, c'est-à-dire- permettez-moi l'expression -dans l'espace de vie ou ou l'espace de régulation des collectivités. Deuxièmement, nous avons interrogé les grandes associations d'élus. L'Assemblée des départements de France a répondu que les départements ne disposaient pas tous des mêmes moyens et que les plus petits pouvaient manquer d'expertise juridique. En bref, l'Assemblée des départements de France a souhaité que les mesures envisagées pour les communes puissent aussi concerner les départements. Nous avons donc substitué au droit à l'erreur des communes, qui figurait dans la rédaction initiale de la proposition de loi, un droit à l'erreur pour l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements. Troisièmement- exercice un peu prétentieux, et je vous prie de m'en excuser -, nous avons essayé non pas de nous immiscer dans votre cerveau, mais d'anticiper vos observations techniques sur le thème « les élus veulent des compétences, mais, c'est toujours pareil, ils n'en acceptent pas les responsabilités ». Rien de tout cela dans le cas précis : pas d'impunité, pas d'irresponsabilité, pas de faveur, vous disais-je. Nous avons scrupuleusement repris les exclusions prévues par le CRPA et dictées par le respect des normes internationales, par le maintien de l'ordre public ou encore par la santé publique. Il nous semble que ce qui était bon en 2018 pourrait le rester en 2020.

quelles situations seraient concrètement concernées par cette extension du droit à l'erreur aux collectivités ». Les collectivités peuvent commettre des erreurs, comme tout le monde, et sont soumises, comme les particuliers ou les entreprises, au droit. Si l'histoire du droit public, qui compte de nombreux spécialistes dans cet hémicycle, est basée sur une lente évolution à partir des prérogatives de puissance publique, les collectivités, dans une forme de convergence juridique, sont de plus en plus soumises aux mêmes règles que les acteurs de droit commun : elles paient la TVA, l'impôt sur les sociétés, des cotisations sociales et sont soumises à de multiples régulations, notamment celles des fameuses autorités administratives indépendantes.

Pourquoi, en d'autres termes, monsieur le secrétaire d'État, dire oui au droit commun en décembre 2019 et dire non en janvier 2020 ? Il est vrai, enfin, que le CRPA ne s'applique pas aux droits dits « spéciaux ». J'ai pu vérifier

de subsidiarité ou de « supplétivité »- je m'excuse de cette formule un peu technocratique, mais qui a l'avantage de reprendre un grand thème, celui de la subsidiarité, commun au Président de la République

vous convaincre. En des temps où la critique est aisée, où la solitude du pouvoir peut être légèrement pesante, acceptez les satisfactions qui vous sont proposées.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, madame, monsieur les auteurs de la proposition de loi, mesdames, messieurs les sénateurs,

et dont il résulte un droit général à la régularisation en cas d'erreur au profit des particuliers et des entreprises, reconnu aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration. Mme la sénatrice Vermeillet, à l'occasion de la discussion de ce projet de loi, avait déposé un amendement tendant à étendre ce droit aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

Ces interrogations demeurent entières aujourd'hui avec cette proposition de loi, puisqu'il apparaît difficile d'identifier les situations dans lesquelles pourrait s'appliquer le droit à l'erreur des collectivités territoriales. Il ne semble en effet pas exister, en l'état actuel du droit, de vide juridique qui ferait peser sur les collectivités locales un risque de préjudice en cas d'erreur commise de bonne foi. Le contrôle de légalité des actes, notamment budgétaires, de rang constitutionnel, prévoit ainsi que les préfectures assurent des missions de conseil et d'appui juridique aux collectivités territoriales, dans le cadre d'une phase gracieuse de dialogue avec les élus. Ces missions des préfectures s'appliquent d'ailleurs, en dehors du contrôle de légalité, à la demande des collectivités territoriales qui auraient des doutes sur le bien-fondé de certaines de leurs

que je suis obligé de constater que les restrictions apportées par la commission des lois, tant pour placer ce texte au sein du seul code général des collectivités territoriales, que vous avez qualifié d'espace de vie ou de régulation des collectivités, que pour sortir

Vous avez rappelé à plusieurs reprises dans votre rapport et en commission que « la vie est aussi faite de symboles ». Il est vrai que, la politique, ce sont aussi des symboles. Cependant, il appartient au Gouvernement de ne pas en rajouter dans la surenchère législative, qui nuit à la lisibilité du droit et à sa compréhension par les collectivités territoriales comme par nos concitoyens.

avec les régimes spécifiques de droit à l'erreur existants, même si la commission des lois a prévu un certain nombre de restrictions. Il est à noter enfin que le texte qui est proposé

ne s'applique qu'en cas de méconnaissance d'une règle applicable ou de commission d'une erreur matérielle pour la première fois. Or la proposition de loi ne reprend pas la notion d'erreur isolée, ce qui la rend applicable en cas d'erreurs matérielles répétées. Le texte est donc potentiellement plus permissif à l'égard des collectivités territoriales que ce que la loi Essoc a prévu pour les usagers et les entreprises.

ou que vous vous souviendrez de Portalis exigeant que la loi ne soit pas trop bavarde, vous ferez votre choix. Quant à moi, je vous suggère de retenir la valeur des symboles. » Permettez au Gouvernement- peut-être le président Bas ajoutera-t-il : « pour une fois » -de rester attaché à la position de Portalis.

force est de constater que le risque pour une collectivité locale de commettre des erreurs et même de voir sa responsabilité engagée s'est accru avec la multiplication des normes et la complexification des procédures administratives à respecter. En effet, les collectivités territoriales sont désormais soumises à des procédures de plus en plus complexes et de plus en plus formalisées, au même titre que certains acteurs économiques. C'est notamment le cas en matière de droit de la fonction publique ou de la commande publique. De surcroît, les collectivités territoriales se retrouvent aussi de plus en plus souvent soumises aux mêmes règles que les acteurs économiques de droit commun. À ce titre, comme les entreprises, elles perçoivent la TVA, paient des cotisations sociales et l'impôt sur les sociétés ou participent au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Cet assujettissement à des règles identiques les confronte aux mêmes acteurs, telles la DGFiP ou les Urssaf, dont elles sont devenues, de fait, des usagers à part entière.

L'objet de la proposition de loi que nous examinons cet après-midi est précisément d'étendre le droit à l'erreur aux communes et établissements publics de coopération intercommunale. Je me félicite que la commission des lois ait décidé de soutenir ce texte, qui reprend majoritairement des dispositions déjà adoptées par le Sénat à l'occasion de l'examen de la loi pour un État au service d'une société de confiance, dite « loi Essoc Confortant le dispositif proposé, elle n'a apporté au texte que des modifications visant à en étendre la portée ou en améliorer l'efficacité. Elle a ainsi tenu à clarifier le champ d'application de la proposition de loi en supprimant le renvoi opéré aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration dans sa rédaction initiale et à créer un droit à l'erreur autonome applicable aux collectivités territoriales. Je me réjouis également que la commission ait élargi le bénéfice de la proposition de loi à l'ensemble des collectivités territoriales et à leurs groupements, et non plus seulement aux communes et à leurs groupements. De plus, je ne peux que me féliciter que la commission ait sécurisé l'articulation entre ce nouveau principe et le droit existant, en prévoyant que le droit spécial ne s'appliquera que s'il a pour objet ou pour effet d'assurer une protection équivalente à celle conférée par le nouveau droit à l'erreur au bénéfice des collectivités territoriales. Enfin, la commission a supprimé la notion de manquement commis pour la première fois, qui trouve difficilement à s'appliquer à des personnes morales de droit public. L'absence de sanction resterait subordonnée à l'absence de fraude ou de manquement délibéré de la part de la collectivité ou du groupement en cause. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, toujours attentif aux préoccupations exprimées par les collectivités territoriales, le groupe Les Indépendants soutient pleinement l'objectif visé par cette proposition de loi. C'est pourquoi l'ensemble de mon groupe votera en faveur de ce texte. Très bien

dans leurs relations avec les administrations et les organismes de sécurité sociale. En tant que cosignataire de la présente proposition de loi, je ne peux naturellement que m'en féliciter. Cette fois, les opposants à cette mesure ne pourront plus, comme cela a été le cas dans le cadre de l'examen de la loi Essoc du 10 août 2018 instituant un droit à l'erreur en faveur des usagers, arguer du fait qu'un tel dispositif n'entre pas dans l'objet de la réforme. Il s'agit là d'un texte autonome dont l'objet est clairement explicité. ne peut valider l'argument d'opposition, avancé dans le cadre de l'examen de la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 et selon lequel l'extension du droit à l'erreur aux collectivités territoriales transformerait ces dernières en usagers de l'administration de l'État. En effet, comme l'a relevé le rapport de notre excellent collègue Philippe Bonnecarrère, un tel argumentaire ne saurait tenir devant l'évidence de notre droit, qui leur reconnaît d'ores et déjà une qualité d'usager à part entière en matière fiscale et sociale. L'article L. 62 du livre des procédures fiscales donne ainsi aux collectivités territoriales et à leurs groupements la possibilité de se prévaloir du droit à la régularisation de leurs erreurs en matière d'impôts, applicable à tout contribuable. En matière sociale, le constat est le même, puisque le décret du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l'erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale semble également assimiler les collectivités territoriales et leurs groupements aux employeurs, au sens du code de la sécurité sociale, notamment lorsqu'elles sont amenées à verser des cotisations sociales. C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'audition effectuée par notre rapporteur de représentants de la direction de la sécurité sociale, qui ont confirmé que l'application des dispositions de ce décret aux collectivités se fondait sur l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne le contrôle des Urssaf et les majorations applicables en cas de redressement. Parce que nos collectivités locales ne cessent de se voir attribuer de nouvelles charges, et ce sans compensation, parce que les lois et règlements ne sont pas toujours aisés à maîtriser, les collectivités, en particulier les petites communes et leurs groupements, souvent isolés et dépourvus de service juridique, doivent aussi pouvoir bénéficier, au même titre que leurs concitoyens, du regard bienveillant de l'État dans les démarches et procédures qu'elles ont à accomplir. D'ailleurs, cette proposition de loi de bon sens conforte la volonté affichée du Gouvernement de redonner confiance à nos élus, comme il l'a manifesté au travers de la loi Engagement et proximité avec l'instauration d'un nouveau rescrit administratif pour sécuriser l'exercice de leurs compétences. Monsieur le secrétaire d'État, nous sommes bien ici dans le domaine du symbole. Si vous voulez vraiment

dont ils bénéficiaient par le passé, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont pas à l'abri d'erreurs et d'omissions. Il est légitime

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, nous commençons à être familiers du concept de droit à l'erreur, mais un bref rappel peut être utile : ce qu'on appelle communément « droit à l'erreur » constitue en réalité un droit à régularisation en cas d'erreur. Pour les citoyens, ce dispositif figure désormais au sein du code des relations entre le public et l'administration. Il ne s'agit pas de consacrer pour les collectivités un droit à l'impunité, un droit à la faveur, comme l'a dit notre rapporteur, un droit à la négligence, à l'incompétence ou un passe-droit Divers projets de loi de simplification, ces dernières années, ont ancré ce principe dans notre droit. Un ancien ministre chargé de ces sujets, M. Thierry Mandon, rappelait cependant, à la fin de 2017, que beaucoup de ces questions ont été monopolisées par Bercy au sein de l'exécutif, et ce quelles que soient les majorités. Cela a eu des avantages : des progrès importants ont été faits en matière de dialogue sur la sphère fiscale. Cela a aussi eu des inconvénients : une vision très, trop centrée autour des questions de finances. La chambre haute, dans sa grande sagesse, avait tenté d'introduire des inflexions à destination des collectivités locales. C'est la genèse de notre débat du jour, qui s'appuie sur l'amendement de notre collègue Vermeillet au projet de loi dit « Société de confiance ». Pour notre collègue, l'extension de ce dispositif de droit à l'erreur aux collectivités repose sur les mêmes principes que ceux qui ont présidé à sa création pour les usagers. Il s'agit d'assurer que les relations entre l'État et ses services, d'un côté, et les collectivités territoriales, de l'autre, soient fondées sur le conseil et l'accompagnement, plutôt que sur le contrôle et la sanction. C'est d'autant plus nécessaire pour les collectivités qui ont des moyens humains et juridiques limités, dans un environnement où les contraintes administratives restent importantes, et ce en dépit des efforts de simplification entrepris depuis plusieurs années.

tournée vers le grand public. Admettons ... Mais cet argument ne tient plus aujourd'hui grâce à cette proposition de loi dédiée. Ensuite, le Gouvernement ne voyait pas du tout quelles situations étaient visées. Mes collègues, notamment Sylvie Vermeillet, ont donc illustré par de nombreux exemples très étayés les situations concernées.

de régler tous les problèmes potentiels. J'ai des doutes sur l'effectivité du contrôle de légalité sur le terrain ; je pense que les sénateurs expérimentés me rejoindront sur ce point. Par ailleurs, le rescrit ne prend pas en considération tous les champs couverts par le droit à l'erreur. Un débat existe sur des limites à apporter à ce droit à l'erreur pour les collectivités. Les grandes collectivités n'en auraient pas besoin. Je ne comprends pas cet argument ! La complexité existe à tous les étages. Si l'on procède par analogie, il faudrait restreindre le droit à l'erreur pour les particuliers sur des critères de ressources ou d'éducation. Cela n'a pour moi guère de sens. A-t-on mis en place des limites pour le droit à l'erreur des plus grandes entreprises ?

depuis 1982, les actes de la décentralisation se succèdent, tous accompagnés de discours bienveillants sur les vertus de l'action locale et des élus. L'acte I a vu la suppression de la tutelle administrative, le transfert du pouvoir exécutif du préfet au président du conseil général et l'instauration du transfert de ressources. visait l'autonomie financière des collectivités territoriales, le transfert de nouvelles compétences et la constitutionnalisation de la région. L'acte III, quant à lui, a consacré l'avènement d'une forme de contractualisation entre l'État et les et les territoires. Il semble ainsi que les gouvernements successifs s'entendent pour présenter ces réformes comme procédant d'une confiance pérenne en l'action territoriale. Notre assemblée ne pourrait que s'en réjouir si les actes suivaient toujours réellement ces discours. Oui, notre assemblée possède par essence une idée claire des réalités locales et a le privilège de porter ici, en connaissance de cause, la voix des territoires Or il est aujourd'hui malheureusement banal de rappeler que les collectivités territoriales peinent à exercer sereinement les compétences qui leur ont été transférées. D'une part, ces transferts ont été nombreux, et ils n'ont pas été accompagnés des moyens nécessaires à leur bon exercice. D'autre part, et c'est l'objet de mon intervention, leur situation est aggravée par la complexification croissante du droit. C'est là encore, hélas, un lieu commun. Ainsi, les textes de simplification du droit pullulent. La récente création d'un droit à l'erreur au profit des usagers de l'administration procède de la même prise de conscience. C'est pourquoi nous avions quasi unanimement défendu au Sénat, pendant la discussion de la loi Essoc, un amendement qui visait à étendre le champ d'application de ce droit à l'erreur aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Rejeté à l'Assemblée nationale par la majorité, nous l'avons porté de nouveau lors de l'examen de la loi Engagement et proximité. Cette demande transcende les clivages partisans, parce qu'elle touche à l'exercice même des compétences de l'élu local, et particulièrement des maires des petites communes, auxquels tant de Français sont attachés. Face à la complexification de notre droit, à la multiplication des procédures, il devient difficile pour les collectivités d'agir sans commettre d'erreurs. Cela est particulièrement vrai pour les plus petites d'entre elles et les EPCI qui ne comptent pas de grande commune en leur sein. Ce manque de moyens les prive de service juridique, d'une expertise approfondie, comme du recours ponctuel à des cabinets spécialisés. Dans un département comme le mien, le Cantal, de nombreuses petites communes sont incapables de faire face à ces évolutions. Comment voulez-vous qu'un secrétaire de mairie, présent une fois par semaine et le plus souvent dépourvu d'une formation juridique appropriée, ne commette jamais la plus petite des erreurs ? Or celle-ci peut être lourde de conséquences, d'autant que le contrôle de légalité des préfectures pâtit, lui aussi, d'un manque de moyens. Il arrive dès lors souvent que des collectivités perdent le bénéfice de subventions dont elles ont besoin en raison d'omissions minimes et involontaires, et il en va ainsi de nombreux actes juridiques. Ces conséquences disproportionnées pénalisent nos collectivités et, partant, nos concitoyens. L'objet de cette proposition de loi est d'y remédier. Le groupe du RDSE la soutiendra, comme les précédents amendements qui allaient en ce sens. Nous demandons non pas de nouveaux moyens, mais simplement que l'État prenne en compte, avec bienveillance, les difficultés que rencontrent les collectivités territoriales. Reconnaître ce droit à l'erreur serait un symbole rassurant et bienvenu de cette considération. Comme je l'ai dit, ce sont surtout les petites communes qui gagneraient à ce que cette proposition de loi soit adoptée. À l'avenir, pourquoi ne pas imaginer, le jour où le droit à la différenciation aura une portée normative effective, de limiter le champ d'application de ce droit à l'erreur aux plus petites collectivités ?

assemblées. La mauvaise foi sur laquelle repose notre droit à l'erreur est l'un de ces mots « caoutchouc » qui abondent dans notre droit positif et qui suscitent des quiproquos sans cesse renaissants

dispose, pour l'essentiel, que la preuve de l'absence de bonne foi doit être rapportée par l'administration, au même titre que pour les manoeuvres frauduleuses. Nous le savons sur ces travées, le droit à l'erreur n'est pas une maigre avancée : c'est une révolution administrative, par l'assouplissement de l'unilatéralité des actes, par l'inversion de la charge de la preuve, par la « subjectivisation »- pardon de ce nouveau mot un peu techno, monsieur le rapporteur -du droit administratif. Encore une fois, le bon sens semble justifier une extension générale de ce droit de régularisation d'erreurs commises de bonne foi par les collectivités territoriales dans leurs relations avec l'État et les organismes de sécurité sociale, fussent-elles coupables de L'inflation normative, le millefeuille administratif et le méli-mélo procédural semblent, en effet, plaider en faveur d'une telle extension. Notre rapporteur a d'ailleurs sécurisé juridiquement cette éventualité par l'apport de quelques rectifications techniques, notamment en autonomisant le droit à l'erreur du code des relations entre le public et l'administration et en élargissant le bénéfice du droit à régularisation à l'ensemble des collectivités territoriales et à leurs groupements. Un certain nombre d'entre nous reste néanmoins sceptique sur l'apport réel, en pratique, de ce texte, les préoccupations formulées par les auteurs de la proposition de loi semblant avoir été partiellement satisfaites par le principe de rescrit préfectoral, institué par la loi Engagement et proximité. Avant d'adopter un acte susceptible d'être déféré, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent ainsi désormais saisir, en amont, le représentant de l'État compétent pour contrôler la légalité de leurs actes. Ce « conseil de légalité », sous forme d'une prise de position formelle, permettra d'accompagner la mise en oeuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leurs exécutifs. les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent déjà se prévaloir du droit général à la régularisation de leurs erreurs en matière fiscale et sociale, puisqu'ils sont assimilables aux employeurs visés par les dispositions du code de la sécurité sociale lorsqu'ils sont amenés à verser des cotisations à travers des dispositions législatives ou réglementaires particulières. Si l'on suit ce raisonnement, dans la pratique concrète, les collectivités territoriales bénéficient aujourd'hui d'un droit à l'erreur.

car l'officialisation du droit à l'erreur n'éteint pas la défiance liée à la complexité des règles à suivre, pas plus qu'elle ne clarifie un processus décisionnel aussi centralisé et normalisé, en raison de la multiplication des normes qui désarme des collectivités sans compétence juridique suffisante. Le droit à l'erreur est, bien sûr, une mesure palliative à l'inflation des normes, qui est notre première préoccupation. La prudence de Portalis trouve tout son écho s'agissant de simplification. Ces réserves étant exprimées, le groupe La République En Marche ne souhaite pas s'opposer ... Ah ! ... à ce que le Sénat pose un acte symbolique

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, il s'agit, comme on le sait, de réintroduire dans la loi un amendement adopté par le Sénat lors

Tout d'abord, parce que ce texte clairement d'affichage était destiné à montrer que le Gouvernement se préoccupe des relations des Français avec l'administration de l'État au sens large, sans un sou supplémentaire, bien sûr, pour permettre à ladite administration de remplir effectivement sa nouvelle mission rendre confiance aux citoyens par la câlinothérapie. Aujourd'hui, l'administration publique n'administre plus : elle donne des conseils et rend des services. Son objectif n'est plus de concilier efficacité et équité de traitement des citoyens, mais de leur donner confiance dans leur administration, donc en eux-mêmes, donc dans leur pays et, accessoirement, dans le Gouvernement. C'est d'abord un service social. Ensuite, parce que ce texte était constitué d'un bric-à-brac de dispositions disparates, sans lien entre elles, voire avec l'objectif poursuivi. Parmi elles, le produit d'appel, objet de la présente proposition de loi : « le droit à l'erreur » pour les personnes de bonne foi ayant méconnu pour la première fois une règle et ayant régularisé leur situation, volontairement ou à la demande de l'administration. une disposition qui ne mange pas de pain, comme on dit chez nous en Provence, mais probablement ailleurs aussi. Pourtant, le Gouvernement avait, lors de l'examen du projet au Sénat, refusé de l'étendre aux collectivités territoriales. Il est vrai que les collectivités territoriales, quoi qu'on en dise, n'occupent pas la même place que les entreprises dans le coeur du Gouvernement.

ce droit à l'erreur se borne à inscrire dans la loi des pratiques existantes qu'un ou plusieurs décrets, voire quelques circulaires auraient suffi à généraliser assez facilement. Voter cette extension d'une disposition de faible portée à l'intérieur d'un texte clairement publicitaire n'étant pas ce que nous préférons, mon groupe, reconnaissant qu'il

Maurey et Sylvie Vermeillet vise à créer un droit à l'erreur des collectivités locales et de leurs groupements dans leurs relations avec les administrations de l'État, ses établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif. Ce texte, porté par le groupe Union Centriste, tente de répondre aux préoccupations qu'un nombre croissant de collectivités territoriales font entendre, en particulier les plus petites d'entre elles, bien sûr, pour lesquelles les moyens sont nécessairement plus limités, mais pas seulement celles-là. Toutes Toutes demeurent en effet, quelle que soit leur taille, de plus en plus soumises aux mêmes règles que les autres acteurs économiques et juridiques, par exemple en matière de procédure fiscale ou de marchés publics, de sorte que c'est bien l'ensemble des collectivités qui sont devenues des usagers à part entière de l'administration. Je tiens ici à saluer l'initiative prise par notre collègue Sylvie Vermeillet, qui, forte de ce constat, fit adopter lors de l'examen au Sénat du projet de loi Essoc un amendement visant à étendre le droit à régularisation aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Cette mesure, quoique soutenue sur l'ensemble des travées de cet hémicycle, n'aura, comme trop souvent, hélas, pas survécu à la navette parlementaire. Reste que la question a eu le mérite d'avoir été posée, et l'occasion nous est aujourd'hui donnée d'apporter une réponse opportune en remettant l'ouvrage sur le métier. J'aimerais revenir sur les arguments pour le moins évasifs avancés alors par le Gouvernement. Il nous avait d'abord été rétorqué que le droit à l'erreur était donné aux usagers de l'administration, et non aux administrations elles-mêmes, de sorte que l'objectif de la réforme en eût été brouillé. Le Gouvernement avait ensuite évoqué un problème de praticabilité, excipant du fait qu'il était concrètement difficile d'identifier les situations qui justifieraient l'élargissement de ce droit en dehors des relations entre les administrations et les usagers. Chacun de ces arguments ne résiste pourtant pas à un examen rigoureux des faits. Je remercie Sylvie Vermeillet d'avoir donné des exemples extrêmement concrets lors de son intervention. Certes, nul ne contestera que les collectivités territoriales une forme d'administration, au sens large du terme, mais cette position d'administration ne saurait être, dans les faits, exclusive de la condition d'usager. À l'instar des entreprises, à qui est reconnu ce droit à régularisation, les collectivités, qui ont une personnalité morale distincte, paient l'impôt sur les sociétés,

On ne voit donc pas très bien en quoi l'application du droit à l'erreur aux collectivités territoriales en diluerait le principe. C'est oublier surtout, et cela a été rappelé en commission des lois, qu'il existe déjà au profit des collectivités territoriales des droits à l'erreur spéciaux en matière fiscale et sociale. À cet égard, la suppression par la commission des lois du renvoi aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et conséquemment la création d'un droit à l'erreur véritablement autonome, permet de distinguer les collectivités du public, à qui s'adresse ce code, et dissipe ainsi toute équivoque. Qu'il me soit ici permis de féliciter le rapporteur de la commission des lois, notre collègue Philippe Bonnecarrère, pour la qualité de son travail et sa sagacité coutumière. Outre l'autonomisation d'un droit à l'erreur dans le code général des collectivités territoriales, nous saluons les clarifications de bon sens apportées à la mouture initiale du texte, en particulier l'ouverture de ce droit nouveau à l'ensemble des catégories de collectivités, en conformité avec ce qu'avait déjà adopté la Haute la Haute Assemblée lors de l'examen du projet de loi Essoc, mais aussi le renforcement de la protection octroyée aux collectivités, de sorte que les dispositions de la proposition de loi ne viennent pas obérer les protections offertes, par ailleurs, par le droit spécial à l'erreur. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, ce texte a été pensé pour entendre, accompagner et écouter les collectivités territoriales dans le cadre des missions qu'elles accomplissent et des procédures qu'elles sont amenées à enclencher au quotidien. Celles-ci appellent, nous le savons tous au Sénat, une ingénierie de plus en plus ardue. Pour que se concrétise cette ambition porteuse à l'égard des élus locaux, dont nous portons la voix, je vous invite à adopter sans réserve la présente proposition de loi. La parole

dite « loi Essoc », a consacré l'introduction dans le code des relations entre le public et l'administration d'un nouveau droit, improprement qualifié de « droit à l'erreur », puisqu'il s'agit d'un droit à régularisation en cas d'erreur. L'article L. 123-1 dudit code prévoit ainsi qu'« une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué Lorsque le Sénat a examiné le projet de loi Essoc, que j'ai eu l'honneur de rapporter avec Jean-Claude Luche pour la commission spéciale, j'étais chargée de ce sujet. En commission, j'avais alors soutenu l'initiative de notre collègue Sylvie Vermeillet visant à étendre le bénéfice du droit à régularisation en cas d'erreur aux collectivités territoriales et à leurs groupements, que je considérais comme fort opportune. Ce dispositif, introduit dans le texte de la commission à l'unanimité, avait été voté par notre assemblée, bien consciente que, tout comme les usagers, les collectivités territoriales et leurs groupements ont aussi besoin du regard bienveillant de l'État et des organismes de sécurité sociale dans le cadre des missions qu'ils doivent accomplir au quotidien et des procédures qu'ils doivent engager dans des conditions parfois difficiles. L'Assemblée nationale avait refusé de reprendre cet apport du Sénat. En commission mixte paritaire, malgré notre proposition de réserver ce droit aux petites collectivités, nous nous étions heurtés à une opposition absolue, au simple motif que cette innovation « ne correspond pas à l'esprit d'un texte dont la préoccupation principale est de simplifier les démarches des usagers de l'administration, qu'ils soient particuliers ou professionnels Je suis donc très satisfaite de voir cette idée revenir grâce à la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Au moins l'argument de ne pas correspondre à l'esprit d'un projet de loi ne pourra plus nous être opposé. Quant à l'autre argument que le Gouvernement avait soulevé, selon lequel il lui paraissait « concrètement difficile de percevoir quelles situations particulières justifieraient l'extension de ce droit en dehors des relations entre les administrations et les usagers opposés », je pense qu'il témoigne surtout d'une grande méconnaissance de ce que vivent les collectivités dans le maquis des réglementations et des formulaires administratifs. Nous le savons tous, le rôle de conseil des préfectures auprès des collectivités territoriales est indispensable, mais les services de l'État n'ont aujourd'hui plus forcément les moyens d'apporter l'appui juridique et l'expertise dont ont cruellement besoin les plus petites communes, souvent démunies face à la complexité et à la multiplicité des procédures. C'est pourquoi je voterai avec conviction cette mesure de bon sens, que la commission des lois a précisée et améliorée en ouvrant ce nouveau droit à l'ensemble des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales. Monsieur le secrétaire d'État, j'ai bien entendu les raisons pour lesquelles vous n'acceptez pas cette proposition de loi.

Autant je suis convaincu de la nécessité d'accompagner plus fortement les collectivités de petite taille en matière d'ingénierie, autant, si nous devions trouver un terrain d'entente sur cette question

puisse, certes, sous l'égide gouvernementale, trouver une issue favorable dans le texte 3D. Concernant l'amendement présenté par M. Maurey, nous comprenons tous son idée : il est important que la preuve de la mauvaise foi reste à la charge de l'administration. Je précise cependant que ce principe me paraît maintenant largement acquis. Il sous-tend l'ensemble des droits spéciaux en cette matière. Vous dire que cette précision est nécessaire serait vraiment excessif. Elle ne nuit pas au texte, sauf à considérer que tout ajout en soi ne fait pas gagner en clarté la disposition. La commission s'en remet donc à

imposant une obligation de demander les pièces manquantes dans un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour l'aide de la DETR et pour la DSIL. En revanche, je reconnais volontiers, tout en émettant un avis défavorable, que la question posée par le président Maurey est pertinente.

qui nous paraît assez éloignée de la réalité du terrain, même si j'entends, comme M. le rapporteur, que des situations peuvent parfois être différentes d'un territoire à un autre. En tout cas, il ne s'agit pas pour nous d'inciter les services

Nous ne souhaitons pas que les préfets refusent une subvention à un projet intéressant au motif d'une simple erreur qui aurait été commise par la commune ou l'EPCI. Je veux aussi préciser que, si l'amendement était adopté, il ne viendrait nullement créer un droit pour l'obtention d'une subvention au profit des projets ainsi régularisés, puisque le préfet reste le maître de la décision d'octroyer la subvention- cela, je crois que nous le partageons -, l'octroi d'une subvention relevant du pouvoir d'appréciation des autorités qui l'attribuent et le bénéfice d'une subvention étant conditionné au respect par le demandeur des critères au-delà même des questions de forme. L'amendement proposé est satisfait- M. le rapporteur l'a dit -par le droit et peut-être de manière indirecte. Le caractère complet du dossier

le dossier est réputé complet au bout d'un délai de trois mois. En cela, votre amendement trouve donc satisfaction. Sur un plan plus général, le droit distingue déjà très bien la vérification de la complétude du dossier et la décision d'attribution elle-même à l'article R. 2334-25 du code général des collectivités territoriales. En effet, il y est précisé que « l'attestation du caractère complet du dossier de même qu'une dérogation accordée sur le fondement du II de l'article R. 2334-24 ne valent pas décision d'octroi de la subvention ». Le droit en vigueur prévoit donc d'ores et déjà une forme de droit à l'erreur en cas de dossier incomplet, même si cela ne se présente pas tout à fait sous la forme que vous proposez dans l'amendement. Enfin, votre amendement- en tout cas, sa présentation -met en avant la complexification des dossiers et la moindre assistance des services de l'État, alors que nous nous efforçons de mettre en oeuvre un mouvement de simplification. Je précise devant vous que les règles de gestion des différentes dotations d'investissement ont été très largement harmonisées, ce qui facilite les demandes de subventions. Elles ont été rassemblées dans une circulaire unique, dont la première édition date de 2019, ce qui nous amènera, je l'espère, à répondre à l'invitation de M. le rapporteur à veiller à une véritable harmonisation et homogénéité des règles d'appréciation

précise que « l'absence d'une pièce au sein d'un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne peut conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante

Je crois que, pour le coup, vous allez absolument dans le sens contraire : vous risquez d'envoyer un signal qui va leur faire très mal ! Notre texte propose simplement d'accorder le droit à l'erreur aux petites communes, comme vous l'accordez déjà aux entreprises du CAC 40. Cela me semble tout à fait légitime. La

territoriales, l'octroi ou le bénéfice d'une subvention relève non du droit mais de l'appréciation par l'autorité délivrant la subvention du respect d'un certain nombre de critères et de la qualité des projets. C'est la raison pour laquelle l'instruction d'un dossier valant obtention d'un droit et l'instruction d'un dossier de demande de subvention

considérer que les collectivités locales sont des sous-traitantes, voire des filiales de l'État. Or nous avons une liberté

Centriste, la discussion de la proposition de loi visant à créer un droit à l'erreur des collectivités locales dans leurs relations avec les administrations et les organismes de sécurité sociale, présentée par

la demande du groupe Union Centriste, la discussion de la proposition de loi relative à la déclaration de naissance auprès de l'officier d'état civil du lieu de résidence des parents, présentée par M. Hervé Marseille et plusieurs de ses collègues

Pour autant, il faut souligner un déséquilibre territorial, puisque près de la quasi-totalité de ces naissances est enregistrée dans seulement 500 communes. Bon nombre de villes et de villages restent vierges au chapitre des naissances, et ce phénomène ne cesse de s'accroître au gré des fermetures des hôpitaux et des maternités. Bien entendu, des futurs parents, des femmes choisissent que l'accouchement se fasse à domicile, mais cette pratique demeure aujourd'hui très marginale en termes de statistiques. La notion même de maison ou de ville natale, si chère aux férus d'histoire et de patrimoine, s'évapore au fil des ans, des siècles. Dans les villes où la maternité a fermé, dans les villages dépourvus de structures, il n'existe pratiquement plus de déclaration de naissance. À Meudon, l'une des plus belles villes d'Île-de-France- ville qui compte plus de 45 000 habitants et dont j'ai été le maire pendant une vingtaine d'années -, il n'existe plus sur le papier de « Naissances à Meudon En effet, le service de maternité ayant fermé il y a quatre ans, les accouchements ont donc lieu dans la ville voisine de Clamart, à l'hôpital Béclère, ou à Sèvres ou encore Les restructurations territoriales de l'offre sanitaire ont déjà eu des répercussions sur les administrés en les obligeant à consulter, à se faire soigner ailleurs que dans la commune où ils habitent. Actuellement, on assiste à un « assèchement » des registres d'état civil. Or nous voudrions que les communes ne soient pas seulement là pour enregistrer des décès. Faire vivre nos communes, c'est aussi faire en sorte de valoriser le dynamisme démographique des territoires, de maintenir des archives communales au bénéfice des généalogistes. Depuis près de vingt ans, de manière récurrente, des collègues parlementaires- que ce soit au Sénat, avec avec Robert Badinter il y a quelques années, ou à l'Assemblée nationale, avec M. Bouillon -, des élus ont milité pour une modification de l'article 55 du code civil. Des questions au Gouvernement ont souvent été posées, des amendements ont été déposés à la faveur de textes régissant les collectivités territoriales, et tout récemment encore : je pense notamment lors de l'examen du projet de loi Engagement et proximité. Des propositions de loi en faveur du lieu de domicile des parents ont bien émergé, mais elles ont été repoussées au motif que la possibilité de domiciles distincts représentait un obstacle juridique. Je pense aussi à la proposition de loi présentée en 2003 par Jean-Marc Pastor, cosignée par Robert Badinter, qui préconisait une procédure de double déclaration des naissances au cas où la naissance n'a pas lieu dans la commune où sont domiciliés les parents.

Il est donc proposé de modifier l'article 55 du code civil, qui, je le rappelle, découle de la loi du 20 novembre 1919 et dispose, dans sa rédaction actuelle, que « les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu

lois, quand une naissance surviendra dans une commune autre que celle du domicile des parents, l'officier d'état civil du lieu de naissance enverra une copie intégrale de l'acte de naissance à son homologue du lieu de domicile des parents, qui la transcrira sur ses registres. En outre, ce dispositif serait d'abord mis en oeuvre à titre expérimental, pour une durée de trois ans. Naturellement, cette nouvelle disposition, si elle est adoptée, obligera certains services municipaux à s'adapter, ou plutôt à mettre à jour leur mode de fonctionnement. Je ne pense pas, néanmoins, que la charge de travail puisse être importante. Ce texte constitue une évolution, pas une révolution. Je sais que le Gouvernement est sensible à cette problématique et je ne mésestime pas les précisions et les améliorations à apporter afin de sécuriser définitivement ce dispositif et, par conséquent, les registres de l'état civil.

et plus de quatre-vingts de nos collègues, répond à une demande régulière des maires, qui souhaitent pouvoir faire vivre l'état civil de leur commune alors que plus aucune naissance n'a lieu sur le territoire

Cette concentration des lieux de déclaration des naissances aboutit au dépeuplement des registres d'état civil des 33 100 communes restantes. La présente proposition de loi tend donc à remédier au dépeuplement des registres des naissances de nombreuses communes.

dans la détermination de l'identité juridique de la personne, le « lieu de déclaration de naissance » au « lieu de naissance ». La commission a également adopté un amendement, déposé par notre collègue Michel Canevet, visant à ajouter le « à la liste des lettres comportant des signes diacritiques qui peuvent être utilisées dans les prénoms inscrits à l'état civil. Malgré ces modifications adoptées la semaine dernière en commission, le dispositif du texte n'était pas pleinement satisfaisant du point de vue juridique.

Il me semble que le dispositif adopté par le Sénat ne doit en aucun cas compliquer la gestion financière qui incombe aux maires des petites communes. Deuxièmement, certains risques pour la fiabilité des registres d'état civil persistaient dans le texte adopté par la commission

Enfin, la rédaction initiale de la proposition de loi pouvait engendrer une certaine confusion en faisant coexister une distinction juridique entre lieu de naissance et lieu de déclaration Malgré les améliorations apportées par la commission, en particulier par la suppression de plusieurs coordinations à l'article 2 du texte initial, nos débats ont montré que cette complexité suscitait de nombreuses questions et était source de confusion. Je souhaiterais donc apporter, à ce stade, une clarification qui me semble nécessaire au vu des échanges que nous avons eus en commission. De fait, remplacer la mention du lieu de naissance, sur les actes de naissance et les documents officiels, par celle du lieu de déclaration de naissance n'est en aucun cas souhaitable. Une telle évolution reviendrait à complexifier considérablement l'état civil et serait un contresens juridique, puisque l'identité de la personne repose sur son lieu de naissance, et non sur celui de la déclaration de naissance. En effet, la création d'une personnalité juridique par l'acte de naissance repose sur le constat de la naissance d'une personne physique à une date et en un lieu donnés. Le lieu de naissance est donc constitutif de l'identité des personnes, et il me semble que l'objet de la présente proposition de loi n'est pas de modifier cet état de fait. En raison de ces difficultés juridiques persistantes et à la suite de nos échanges avec le Gouvernement, il nous a donc paru préférable d'adopter le dispositif prévu au travers de l'amendement n° 3, que j'ai déposé au nom de la commission.

L'amendement est le fruit d'échanges avec la Chancellerie ; M. le secrétaire d'État devrait nous confirmer l'accord du Gouvernement sur le dispositif proposé. Cette rédaction permettrait d'expérimenter, pour une durée de trois ans, les registres d'actes dits « miroirs ». Cela répondrait aux difficultés juridiques soulevées plus tôt. Premièrement, le coût pour les communes concernées fera, au même titre que l'ensemble des impacts, l'objet d'une évaluation précise remise au Parlement six mois avant le terme de l'expérimentation. Deuxièmement, Deuxièmement, les éventuelles difficultés en matière de fiabilité des registres d'état civil seront traitées par le biais d'un décret en Conseil d'État. En effet, le fonctionnement du dispositif serait le suivant : les conditions de déclaration d'une naissance, dont le lieu, ne seraient pas modifiées après avoir dressé l'acte de naissance, l'officier d'état civil du lieu de naissance en enverrait une copie intégrale à l'officier d'état civil du lieu de domicile du ou des parents ; si les domiciles des parents sont distincts, une copie intégrale serait envoyée à l'officier d'état civil de chacun des lieux de domicile enfin, les officiers d'état civil concernés seraient tenus non seulement de transcrire la copie d'acte sur leurs registres de naissance, mais également de les tenir à jour afin de pouvoir en délivrer des copies et extraits. En résumé, le lieu de déclaration de la naissance et le lieu de naissance resteraient identiques, à l'image de ce qui est pratiqué aujourd'hui. En revanche, le service public que représente l'état civil des petites communes serait revivifié, ce qui représente, à l'heure où la proximité des services publics fait l'objet de débats nourris, un avantage indéniable pour les citoyens. Par ailleurs, le poids symbolique d'un registre des naissances vide pour les maires de petites communes disparaîtrait, puisque les actes de naissance d'enfants de foyers installés dans leur commune, mais nés sur le territoire d'une autre commune, seraient dorénavant transcrits sur leur registre des naissances. L'expérimentation proposée permettra, à tout le moins, de lever les ambiguïtés sur ce sujet qui revient de manière lancinante nourrir nos débats. Je précise enfin que l'arrêté du garde des sceaux fixant la liste des communes retenues pour cette expérimentation serait pris en

et partagé par tous. La vitalité d'une commune se mesure à l'implication de ses résidents dans la vie et le développement de la communauté, à son nombre d'habitants, au développement de ses infrastructures, à son accessibilité, à son taux d'activité, et à bien d'autres critères Je ne peux ignorer l'attachement des Français à la tenue des registres des naissances ayant lieu sur le territoire de leur commune, qui est l'un de ces critères. L'Insee publie d'ailleurs chaque année des statistiques de naissances par commune-

de l'état civil et emportent des conséquences pratiques importantes pour l'ensemble des communes et villages de France. Il s'agirait en effet d'imposer aux communes de domicile des parents d'établir des actes de naissance pour des naissances ayant eu lieu dans une autre commune. Ces communes de domicile auront donc la charge de mettre à jour les actes ainsi établis à chaque événement nouveau. Un mariage, la conclusion d'un pacte civil de solidarité, un divorce, un changement de nom, de prénom ou de sexe, bien d'autres tous doivent être mentionnés en marge de l'acte de naissance. Ces communes seront ainsi contraintes de recruter et de former des agents à ces nouvelles fonctions d'établissement et de mise à jour des registres de l'état civil. Elles devront également engager des dépenses

ces dispositions me paraissent accentuer le risque de fraude documentaire. En effet, elles dérogeraient au principe général selon lequel les actes de l'état civil doivent être dressés au lieu de l'événement qu'ils relatent, ce qui garantit leur caractère authentique. Cette dérogation irait à l'encontre des objectifs et des dispositifs de fiabilité et de sécurité des actes de l'état civil et des titres d'identité établis sur la base des actes de naissance. Or ces dispositifs sont mis en oeuvre depuis quelques années déjà par les communes de naissance. Permettre à l'ensemble des communes françaises d'établir des actes de naissance constituerait, sur ce point, un recul massif dans la lutte contre la fraude documentaire. Toutefois, comme je vous le disais au début de mon intervention, le Gouvernement est sensible à la demande formulée. C'est pourquoi une évolution des dispositions en vigueur est parfaitement envisageable. Elle devra tenir compte des conséquences financières et juridiques que je viens d'exposer.

conforme à l'article 37-1 de la Constitution, ouvrant la possibilité, pour la ou les communes de domicile des parents, de transcrire sur leurs registres de l'état civil l'acte de naissance établi par la commune de naissance. L'amendement n° 3 que vous examinerez tout à l'heure, qui reçoit l'avis favorable du Gouvernement, vise à appliquer aux actes de naissance les dispositions de l'article 80 du code civil d'ores et déjà prévues pour les actes de décès. Ainsi, l'officier de l'état civil du lieu de naissance établirait l'acte de naissance de l'enfant au vu du certificat d'accouchement et des éléments d'identité du ou des parents cet officier de l'état civil transmettrait sans délai une copie intégrale de l'acte de naissance à l'officier de l'état civil du lieu de domicile du ou des parents ; enfin, ce dernier transcrirait l'acte de naissance sur les registres de l'état civil de sa commune.

viendrait fixer les modalités d'application de cette disposition, en particulier les conditions dans lesquelles celles-ci garantissent la fiabilité et la préservation de l'intégrité des données de l'état civil des personnes intéressées.

Cette proposition d'expérimentation apparaît indispensable pour mesurer les effets de l'introduction de telles dispositions sur les communes, d'une part, et sur la sécurité et la fiabilité des registres de l'état civil,

En effet, introduire l'utilisation d'un ou de plusieurs signes diacritiques régionaux dans les actes de naissance aurait nécessairement une incidence sur l'ensemble des actes et démarches effectués tout au long de la vie des intéressés affiliation à la sécurité sociale, délivrance des titres d'identité, inscriptions scolaires, conclusion de contrats de travail ou de baux d'habitation, établissement d'actes notariés, etc. Pour les communes, une adaptation des logiciels métiers sera nécessaire, ainsi qu'un renouvellement des claviers d'ordinateur et une mise à jour des actes de l'état civil, des titres d'identité, des documents de sécurité sociale et des actes notariés ... Ces implications sont particulièrement larges et, en l'état, et, en l'état, n'ont pas toutes été anticipées. La question de l'admission du tilde dans les actes de naissance, et non dans les actes de mariage ou de décès, peut également se poser.

de ces raisons que le Gouvernement étudie actuellement la faisabilité d'une intégration de certains signes diacritiques pour permettre la prise en compte de l'orthographe de certains prénoms issus de langues régionales. Pour l'heure, le Gouvernement est réservé sur cette disposition.

avant tout à saluer l'initiative du président de notre groupe, Hervé Marseille, qui nous permet de débattre aujourd'hui d'un texte relatif à la déclaration de naissance auprès de l'officier d'état civil du lieu de résidence des parents.

Il s'agit donc d'ouvrir une nouvelle possibilité, et non de créer une obligation. Il n'est nullement question de modifier le lieu de naissance, qui reste attesté par le certificat délivré par la maternité. Avant de revenir sur les fondements de cette proposition de loi, force est de constater que l'idée d'une déclaration de naissance au lieu du domicile avait été avancée au Sénat dès 1999 par des parlementaires de tous bords, mais sans faire l'objet d'une discussion en séance publique. Nos collègues députés ont également été nombreux, au cours des dernières années, à déposer des propositions de loi sur ce sujet sur le bureau de l'Assemblée nationale. Comme cela a été rappelé, ce texte tend à répondre à un problème souligné de manière récurrente par les maires des petites communes, notamment rurales,

de celle-ci. À titre d'illustration, en 2016, 99,6 % des naissances ont été enregistrées dans seulement 500 communes de notre pays. Ce constat n'est pas sans poser quelques difficultés pour les élus locaux et les citoyens.

La concentration des naissances met à mal l'attachement de nos concitoyens à leur commune de domicile. En outre, pour les maires et leurs adjoints, ce dépeuplement des registres de naissance est un signal négatif pour la revitalisation des petites communes et peut être perçu comme non représentatif de la démographie réelle

Vous l'aurez compris, mes chers collègues, afin de limiter ces effets négatifs, la présente proposition de loi tend à laisser aux parents le choix du lieu de déclaration de la naissance de leur enfant. Ils pourraient ainsi déclarer celle-ci au lieu de naissance, comme c'est le cas aujourd'hui, ou au lieu du domicile de l'un d'eux. Par ailleurs, le délai pour effectuer cette déclaration serait porté à huit jours. Je tiens à saluer le travail effectué par notre rapporteur, Agnès Canayer, qui a parfaitement compris l'intérêt et l'enjeu,

Admis dans la langue française depuis l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, le tilde est peu à peu tombé en désuétude et n'est aujourd'hui mentionné dans aucune disposition réglementaire.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, il est rare qu'une niche parlementaire suscite autant d'intérêt à l'extérieur de notre hémicycle ! Je tiens à remercier ici les instigateurs de ce débat

civil de la commune de résidence des parents ne sera qu'optionnelle : elle ne vient donc pas « supprimer le lieu de naissance », comme un journal parisien a pu le titrer ce matin. Des dispositions sont prévues pour prendre en compte le cas de parents séparés. Nos collègues ont rappelé en commission des lois les différences qui pouvaient exister avec le modèle suisse. Je remercie Jean-Pierre Sueur, pertinent comme toujours, d'avoir évoqué le sujet du décès, qui pourrait entraîner les mêmes questions En 2016, 594 000 personnes sont décédées en France : 59 % dans un établissement de santé, 26 % à domicile, 14 % en maison de retraite et 1 % sur la voie publique. Certes, ce dernier point nous fait perdre de vue l'intérêt de notre démarche en matière d'attractivité des petites communes ! Mais si je suis convaincu de l'importance symbolique de cette initiative pour le monde rural, je doute en qu'elle permette de compenser les fermetures de maternités. Notre collègue Jacques Bigot a déposé un amendement visant à s'assurer de l'engagement de l'État pour éviter que des effets pervers n'abîment notre si précieux état civil. La rigueur en la matière est de mise, on le sait.

Nous comprenons que la majorité sénatoriale a choisi une autre voie avec cette expérimentation qui ne nous semble pas totalement sécurisante. Nous ne nous opposerons cependant pas à ces solutions, par souci de compromis, mais l'investissement du Gouvernement pour sécuriser le dispositif retenu est d'une importance capitale.

un risque de discrimination sociale. Ces arguments ne peuvent être balayés d'un revers de la main, mais notre groupe a majoritairement choisi de soutenir ce texte. Nous ne pinaillerons pas.

La commune n'est pas le monde d'hier, le maire est aujourd'hui plus que jamais un acteur essentiel de la République. [ ...] Lorsque le temps du dialogue est venu, c'est d'abord autour de la mairie, autour des maires que les citoyens se sont rassemblés et se sont mis à échanger. Je suis heureux de constater que la proposition de loi de notre collègue Hervé Marseille, que j'ai cosignée, a été adoptée à l'unanimité par la commission des lois, dont je salue le travail, ainsi que celui de la rapporteure, Agnès Canayer. Toutefois, à la lecture du compte rendu des travaux de la commission,

dans chaque commune, une table alphabétique des actes de l'état civil pour les naissances dans la commune, mais également pour les naissances dans une autre commune d'enfants dont les parents sont domiciliés dans la commune.

une quelconque forme de reconnaissance financière. Je rappelle que l'établissement des tables annuelles de l'état civil n'autorise pas la commune de résidence à délivrer une copie ou un extrait d'acte de naissance à la personne intéressée, qui doit donc, toute sa vie, s'adresser à sa commune de naissance. À l'inverse, en ce qui concerne les actes de décès, toutes les communes sont tenues de les établir ou de les transcrire dans le cas où le décès de leur administré est survenu hors de la commune. Cette inégalité de traitement d'état civil a conduit notre collègue Hervé Marseille à faire ce triste constat : « On ne parle plus que des morts dans les villages. Il n'y a plus de naissances. Tout le monde naît dans l'une des 500 maternités et il y

je rappelle que 50 % des communes françaises comptent moins de 500 habitants -à celui d'un officier d'état civil n'établissant plus que des actes de décès et, très rarement, des actes de mariage. Je partage le constat de la commission sur les effets pervers de la concentration des naissances,

Cet état civil laïcisé, nous le devons au décret du 20 septembre 1792. À l'époque déjà, la question de la proximité entre la naissance- l'acte événement -et la déclaration- l'acte document -animait les débats. Par nécessité sans doute, l'enregistrement de l'état civil auprès des municipalités avait été pensé pour satisfaire un besoin pratique : identifier les citoyens en recourant à ceux qui étaient le plus à même de le faire au sein de villages où « tout le monde se connaissait Nous sommes appelés à légiférer sur un dispositif qui, au fond, s'inscrit dans cette symbolique historique un peu mythifiée.

il est proposé de permettre aux parents qui le souhaiteront de déclarer la naissance d'un enfant dans la commune de domiciliation de l'un d'eux. Ce caractère optionnel n'enlève rien à la forte dimension symbolique

Notre groupe était néanmoins réservé quant à l'opportunité d'introduire des dispositions dont la plus-value est peu évidente et les implications concrètes incertaines.

loi : maintenir la mention du lieu effectif de naissance sa transcription dans le registre de l'état civil, à côté de celle du lieu de résidence des parents. L'expérimentation de tels registres d'actes « miroirs », par analogie avec les actes de décès, conduirait l'officier d'état civil du lieu de naissance à établir l'acte original et à en adresser, dans les plus brefs délais, une copie à l'officier de l'état civil du lieu de domicile des parents, qui la transcrirait immédiatement sur ses registres.

La méthode expérimentale, quant à elle, est le bon vecteur pour évaluer, à terme, les effets opérationnels de ce dispositif sur la gestion de l'état civil.

Dans nos territoires ultramarins, les maternités ont souvent été regroupées pour des raisons matérielles. À Mayotte par exemple, trois quarts des 10 000 naissances annuelles sur l'île sont enregistrées au seul centre hospitalier de Mamoudzou, alors que les familles sont disséminées sur l'ensemble des dix-sept communes. La réalité démographique de l'île s'en trouve en quelque sorte faussée. Je me félicite que les dispositions de cette proposition de loi, dont je tiens à remercier les auteurs, viennent corriger cet état de fait.

alors que le risque d'amoindrir la lisibilité actuelle de la réglementation en matière d'inscription des naissances à l'état civil n'est pas négligeable, surtout si, contrairement à ce que j'avais cru comprendre, la mise en oeuvre du nouveau dispositif est précédée d'une période d'expérimentation,

Ce n'est pas un hasard. Il ne reste guère plus de 500 maternités dans notre pays. La conséquence mathématique en est que la quasi-totalité des naissances en France ont aujourd'hui lieu dans moins de 500 communes. Ainsi, les déclarations des naissances ayant lieu sur notre territoire sont concentrées dans à peine plus de 500 registres d'état civil. Il est de moins en moins fréquent qu'une mère accouche dans sa commune de résidence,

que nous examinons cet après-midi permettrait aux parents qui le souhaiteraient de déclarer la naissance d'un enfant dans la commune d'attache de la famille. Il ne s'agit pas de déclarer un autre lieu de naissance : un enfant né au centre

prévoit pas le cas où les parents ne parviendraient pas à s'accorder sur le lieu de domicile ; à cet égard, un risque contentieux existe. Les dispositions de cette proposition de loi pourraient également poser problème en matière de fiabilité des registres. En effet, si une personne décidait de déclarer son enfant au lieu de naissance, puis à son lieu de domicile, les deux officiers d'état civil concernés

amendement précise la procédure en cas de désaccord des parents sur le lieu de déclaration. De même, je me réjouis de la suppression de plusieurs mesures de coordination figurant à l'article 2, pour maintenir dans certains articles du code civil la notion de lieu de naissance. C'est bien le lieu de naissance- et non celui de la déclaration -qui contribue à définir l'identité juridique de la personne. Enfin, je me félicite tout particulièrement de la précision apportée au droit concernant les lettres et les signes diacritiques que peuvent comporter les prénoms inscrits à l'état civil. Nous avons tous en tête l'affaire du petit Fañch : il aura fallu une bataille judiciaire de plus de deux ans pour que la licéité de ce prénom breton

de vous remercier,

L'article 55 du code civil, qui découle de la loi du 20 novembre 1919, dispose que « les déclarations de naissance seront faites, dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu de naissance Cette disposition se justifie précisément en raison de l'ancienneté de cette loi et des pratiques de l'époque. En effet, au début du XX siècle, l'usage voulait que les femmes accouchent à domicile. Au fil des ans, les accouchements se sont déplacés d'abord dans des petites maternités peu éloignées du lieu de résidence, pour ne plus se dérouler de nos jours, à quelques exceptions près, que dans de grands ensembles hospitaliers, localisés dans des villes de plus grande importance. L'exemple de l'hôpital transfrontalier franco-espagnol de Cerdagne s'inscrit parfaitement dans la problématique soulevée par cette proposition de loi. Cet établissement se situe sur le territoire espagnol, à un kilomètre de la frontière française de Bourg-Madame, dans les Sans revenir sur les étapes de sa mise en place, je rappellerai simplement qu'il a fait l'objet d'une déclaration d'intention commune lors du sommet franco-espagnol de Barcelone en 2005, en présence des deux Premiers ministres de l'époque. Cette déclaration s'appuyait sur le traité de Bayonne du 10 mars 1995, qui a posé les bases d'une coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales françaises et espagnoles. européenne a consacré ce projet en apportant plus de 18 millions d'euros, soit 60 % du financement. Sa mise en oeuvre juridique,

Ce GECT définit un périmètre incluant deux cantons français et une comarque catalane. Je ne reviendrai pas sur les difficultés d'harmonisation des législations française et espagnole dans le domaine des pratiques médicales et du droit social qui ont pu être surmontées.

dans le cadre du sommet franco-espagnol de Saragosse du 25 juin 2008. Un accord approuvé le 20 février 2017 à Malaga permet le transport des corps

et la proposition de loi que j'avais déposée à l'Assemblée nationale, à résoudre le problème posé par la naissance d'une centaine de bébés français à l'hôpital de Cerdagne. En effet, ces bébés français font l'objet d'une déclaration au consulat de Barcelone et sont, de ce fait, considérés comme nés à l'étranger et inscrits au fichier du service central de l'état civil de Nantes. Cet organisme public déconcentré dépend du ministère des affaires étrangères ; il délivre les actes de naissance pour les enfants nés à l'étranger Le territoire de compétence du GECT comprend une quarantaine de communes de montagne françaises. Ces bébés devraient donc être enregistrés dans la commune de résidence des parents, ainsi que le prévoit la proposition de loi de mon collègue Hervé Marseille. de mon collègue Hervé Marseille. Au fond, grâce à l'Europe, nous avons pu apporter aux habitants de ces communes de montagne une offre de soins de qualité, en permettant que les futures mères puissent accoucher à proximité de leur commune de résidence, au lieu de devoir faire cent kilomètres sur des routes souvent enneigées ou accidentées.

Cet établissement hospitalier a une vocation européenne. Les frontières administratives doivent être assouplies pour nos concitoyens. On doit privilégier le critère de proximité et considérer le lieu de résidence des parents, comme le rappelle très justement la

de l'état civil à Nantes, mais auprès des communes de résidence des parents. De plus, cette évolution permettrait aux historiens et généalogistes

Il vise aussi et surtout à inscrire, à l'article 79-1 du code civil, que les parents peuvent indiquer les noms et prénoms qu'ils souhaitent donner à l'enfant.

En droit positif, lorsqu'un enfant décède avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, le code civil distingue deux cas. Si l'enfant est né vivant et viable, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance, ainsi qu'un acte de décès.

Par votre amendement, vous entendez définir les critères de viabilité par référence aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. En définissant la viabilité sur le fondement de critères médicaux, l'adjonction proposée à l'article 79-1 du code civil revient en réalité à subordonner l'accès à la personnalité juridique à des critères purement anatomiques. Outre que l'insertion de tels critères médicaux n'a pas sa place dans le code civil, la détermination au niveau législatif de la viabilité emporte des incidences sur le statut du foetus de

interruptions de grossesse pratiquées pour motif médical à un stade tardif de la grossesse, voire aux interruptions volontaires de grossesse. En permettant aux parents de donner un nom à l'enfant sans vie, votre amendement remettre en cause les principes de droit qui régissent la personnalité juridique. En droit français, le nom et la filiation constituent des attributs de cette personnalité. Celle-ci résulte du fait d'être né vivant et viable et ne peut en conséquence être conférée à l'enfant sans vie. Octroyer un nom de famille à l'enfant qui n'est pas né vivant ni viable reviendrait à lui reconnaître la personnalité juridique, ce qui conduirait inévitablement à une modification du statut du foetus, question qui excède, je le répète, l'objet de la présente Le dispositif d'établissement des actes d'enfant sans vie procède d'un équilibre délicat, sensible, entre, d'une part, la douleur des parents confrontés à la naissance d'un enfant sans vie et la reconnaissance symbolique du lien qui les unit à celui-ci, et, d'autre part, nos principes de droit concernant la personnalité juridique. Permettez-moi enfin de rappeler que le décret du 20 août 2008